La séance est reprise.

Républicains. Monsieur le Premier ministre, le sujet est très sérieux, mais votre légèreté à le traiter m'amène à vous proposer une charade. Mon premier est une commune de Loire-Atlantique. Mon deuxième est le résultat d'un fiasco politique du quinquennat précédent. Mon troisième est une zone de 1 600 hectares où les forces de l'ordre républicaines ont été interdites de circuler. Et pourtant, le facteur y portait le courrier des zadistes en droit de toucher les aides sociales Mon quatrième est une zone où le droit de propriété est bafoué par des zadistes construisant des abris en toute illégalité. Mon tout est une zone de non-droit où nos forces de l'ordre sont attaquées alors qu'elles accomplissent avec courage leur mission au nom de l'État. Les Français sont choqués ; les Français sont exaspérés ! Monsieur le Premier ministre, je pense que vous avez compris de quoi je parle ! Comptez-vous réellement rétablir l'ordre public à Notre-Dame-des-Landes ?

Les occupations illégales auxquelles nous mettons un terme en ce moment n'ont pas commencé avec la nomination de ce gouvernement. Elles n'ont pas commencé, monsieur le sénateur- puisque vous avez procédé par charade, permettez-moi d'inverser le questionnement -, avec le quinquennat précédent

C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui va se passer ! Notre objectif, depuis le début de l'opération- celle-ci est placée sous le commandement du directeur général de la gendarmerie nationale et de la préfète, et suivie quotidiennement par le ministre d'État, ministre de l'intérieur, et par moi-même -, est bien de faire en sorte que la liberté de circulation soit rétablie sur les axes qui traversent la zone, et que l'ensemble de ceux qui occupent sans titre et de façon illégale

Et c'est ce que nous faisons ! Vingt-neuf constructions illégales ont été détruites ; elles sont en voie de déblaiement. Nous sommes en train de retirer, benne après benne- elles sont plusieurs dizaines, ces bennes -, des matériaux de construction illégalement installés, stockés et utilisés sur les zones. Vendredi dernier, avec le ministre d'État, ministre de l'intérieur, je me suis rendu sur la commune de Saint-Étienne-de-Montluc pour rencontrer les gendarmes, les pompiers, les membres du parquet de Nantes et de Saint-Nazaire, qui concourent aux opérations avec un professionnalisme exemplaires, face à des provocations que vous connaissez- je le pense -parfaitement. Face aux pressions, ils gardent leur calme. Ils ont subi beaucoup d'assauts.

à ceux des occupants illégaux qui, peut-être, n'auraient pas compris la détermination dudit gouvernement : soit ils entraient dans un processus de respect de la loi, soit ils en tireraient les conséquences et seraient exclus des parcelles qu'ils occupent illégalement. C'est très exactement ce que nous avons dit, monsieur le sénateur, et c'est très exactement ce que nous allons faire. Nous allons le faire avec le souci d'éviter les incidents. Nous allons le faire avec le souci de permettre aux gendarmes de remplir leur mission dans des conditions de sécurité maximale. Mais nous allons le faire, monsieur le sénateur, sans charade, sans légèreté, avec une immense détermination, avec une force tranquille dont je ne voudrais pas que vous puissiez douter le début du commencement d'une seconde. La parole

insupportable aussi, votre façon de gérer l'évacuation, avec 2 500 gendarmes bridés face à 150 zadistes. Vous vous félicitez du démantèlement de 29 squats ; 29 sur 99 au total ... Cela revient à féliciter un élève avec une note de 7 sur 20

Union Centriste. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Monsieur le ministre, M. le Président de la République s'est adressé mardi aux députés européens. Dans la lignée des discours d'Athènes et de La Sorbonne, il a réaffirmé son engagement et sa foi en l'Europe, une Europe démocratique, souveraine, protectrice. Cette Europe renouvelée, une « Europe-puissance » que nous appelons de nos voeux, est aussi confrontée aux replis démocratiques et aux égoïsmes nationaux. Nous pensons que c'est précisément la souveraineté européenne qui doit nous permettre de défendre notre singularité culturelle, nos libertés, notre protection sociale, en même temps que la paix et la stabilité internationale. Pour autant, aujourd'hui, l'Europe politique semble figée. Le dernier Conseil européen l'a montré. Elle a du mal à décider. Les élections se succèdent, à l'issue desquelles les coalitions contraignent, les extrêmes empêchent et un grand nombre de partis traditionnels hésitent. Chacun en convient : l'immobilisme n'est plus une option. Les événements s'accélèrent, le monde change. La France est dans son rôle d'initiatrice de l'intégration européenne. Elle avance des idées nouvelles. Nous voulons améliorer la zone euro, mettre en commun nos moyens financiers, réagir aux pulsions protectionnistes, protéger nos pépites technologiques, bâtir une politique d'immigration commune, nous doter de moyens militaires crédibilisant une posture diplomatique commune. L'heure n'est plus au repli ni au sommeil. Les Européens doivent maintenant démontrer qu'ils sont capables d'affronter ensemble les vrais défis du présent qui conditionnent l'Europe de demain : immigration, sécurité, gouvernance démocratique. Le Président de la République rencontre aujourd'hui la chancelière Merkel. La France et l'Allemagne doivent montrer l'exemple et annoncer une feuille de route Il existe, vous le savez, quelques interrogations sur cette volonté commune de progresser. Quels moyens la France se donne-t-elle pour convaincre ses partenaires européens de la suivre dans ses projets de refondation de l'Europe ? La parole

rêve européen que, je le sais, vous partagez. Le meilleur moyen de mettre un terme à ces vents mauvais est de repartir des fondations de la maison commune. Or les fondations de la maison commune, ce sont les peuples d'Europe ! C'est le sens des consultations citoyennes lancées par le Président de la République à Épinal.

Le coût suivra évidemment un tel rythme. À l'heure où le débat sur la fin de vie et l'euthanasie refait surface, ne serait-il pas essentiel de s'intéresser au bien-vieillir en France ?

Il faudra financer ce cinquième risque. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés ! Seule la solidarité collective peut y pourvoir. Pour appréhender l'enjeu financier des décennies à venir, vous avez évoqué, madame la ministre, l'instauration ministre, l'instauration d'un deuxième jour travaillé non payé, sur le modèle du lundi de Pentecôte. Pour chacun, cela représenterait par jour travaillé un effort de deux minutes. telle mesure apporterait près de 3 milliards d'euros de recettes et contribuerait ainsi à résoudre la crise actuelle. Elle permettrait un accueil dans la dignité des personnes dépendantes. la ministre, ma question est la suivante : cette contribution de solidarité collective, qui résoudra dans un premier temps la crise actuelle, consacrera-t-elle de manière définitive le cinquième risque ? La parole

il convient d'améliorer les conditions actuelles de prise en charge, que ce soit en EHPAD ou à domicile. Nous avons déjà eu de nombreux débats sur le sujet. Nous savons qu'il nous faut trouver de nouvelles pistes pour l'avenir. C'est un impératif de solidarité vis-à-vis non seulement des personnes âgées, mais également des familles. Nous serons tous amenés à profiter de cette solidarité. J'ai effectivement évoqué différentes pistes. Le Président de la République a repris celle de la journée de solidarité ; c'en est une parmi d'autres. Je pense qu'il faudra un large débat sur le sujet. La première étape est d'abord de savoir quel projet de société nous faisons pour accompagner les personnes âgées dépendantes à l'avenir. Aujourd'hui, le modèle domicile-EHPAD est probablement insuffisant et réducteur. Une fois que nous connaîtrons les moyens, nous devrons discuter du financement. Je le rappelle, la journée de solidarité a été voulue par Jean-Pierre Raffarin, et mise en place en 2004. Elle a donné des moyens aux établissements comme

fortune ? ... nous y avons pensé aussi pour les aidants. Si nous y pensons pour les aidants, cela peut aussi se justifier pour les personnes âgées dépendantes : ce sont les mêmes fondements. Nous aurons à y travailler tous ensemble dans les mois qui viennent. Le sujet doit être examiné. Il nécessite un temps de concertation. La parole

Pourtant, nous connaissons encore tous des communes que vous n'avez pas retenues alors qu'elles sont les seules au milieu d'autres communes classées. C'est le cas de Saint-Christophe-de-Double en Gironde. Vous indiquiez ici indiquiez ici que cette carte était « la base de travail pour entamer les discussions avec la Commission européenne », notamment en ce qui concerne « l'application d'un critère de continuité territoriale qui pourrait permettre à certaines communes de réintégrer le zonage Mais la Commission européenne est-elle vraiment ouverte à la discussion ? Merci de nous le dire ! Faisons par ailleurs le calcul. À l'échelon national, force est de constater que les communes classées et les éleveurs bénéficiaires sont en hausse. Ce n'est pas le cas dans certains départements. Ainsi, en 241 éleveurs répartis dans 165 communes étaient classés en ZDS. Avec la nouvelle carte- elle a, certes, des mérites, notamment celui d'introduire des territoires comme le Bazadais, le Coutradais, la pointe du Médoc ou le Blanquefortais -, ce sont seulement 183 éleveurs qui bénéficieront de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels. Il s'agit donc d'acter le retrait de ces aides à 58 éleveurs. Que sera l'avenir de ces exploitations ? Ce sont en moyenne 5 800 euros par an que ne percevront plus ces agriculteurs ; pour certains, cela ira jusqu'à 10 000 euros Vous vous êtes engagé ici à lancer un grand plan d'investissement et à définir de nouvelles mesures avec les professionnels et les collectivités, en particulier les conseils régionaux. Mais ces derniers n'ont plus les moyens d'assumer des compétences nouvelles sans compensation de la part de l'État ! Alors, monsieur le ministre,

nous savions- c'était une demande expresse de la Cour des comptes européenne -qu'il nous fallait modifier cette cartographie pour prendre en compte des évolutions réglementaires, statistiques ou géographiques,

vous l'avez souligné, en macro, ce sont 14 133 communes, et donc autant d'agriculteurs dans chacune de ces communes, qui vont pouvoir bénéficier dorénavant du dispositif des ICHN et de tous les dispositifs d'aides territorialisées, alors qu'il n'y avait que 10 429 communes. Mais vous avez raison d'évoquer la situation particulière de celles et ceux qui sortent de la cartographie. S'il y a effectivement près d'un tiers de bénéficiaires supplémentaires, des communes en sortent. Vous

chaque agriculteur et chaque exploitation fassent l'objet d'un accompagnement spécifique de la part des autorités de son ministère. Il faut que la sortie se fasse en tuilage et que nous puissions mettre en parallèle des dispositifs pour

Permettez-moi d'abord d'apporter, au nom du groupe CRCE, notre soutien plein et entier aux cheminots, aux étudiants et à tous ceux qui défilent cet après-midi pour défendre l'idée qu'ils se font du service public, patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ma question s'adresse conjointement au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Monsieur le ministre d'État, j'imagine votre désarroi en constatant le faible intérêt du Président de la République pour l'agriculture et l'écologie. Curieusement, lors de ses interventions récentes, il a essentiellement évoqué le sujet pour discréditer l'idée d'un nouveau mode de production alternatif et collectif ... Oh ! ... qui germe notamment sur les terres préservées de Notre-Dame-des-Landes. C'est le comble ! Nous ne pouvons plus nous permettre de mépriser les tentatives de ceux qui osent un changement radical. La renégociation de la PAC 2021-2027 est une occasion pour le Gouvernement de prendre ce virage. Le calendrier s'accélère. Lundi, à l'occasion du conseil des ministres européens de l'agriculture, la plateforme « Pour une autre PAC et ses partenaires d'outre-Rhin ont remis leurs propositions communes aux ministres français et allemands de l'agriculture et de l'environnement. Dans six semaines, les grandes lignes de la PAC qui engageront l'Union européenne jusqu'en 2027 seront fixées. Or nous n'avons à ce jour que peu d'informations, même sur la position française, si ce n'est le bruit d'une baisse impensable des crédits de 3 milliards d'euros. Le Sénat s'en est ému le 12 avril en adoptant une proposition de résolution européenne demandant au Gouvernement de défendre une PAC plus ambitieuse que le dernier exercice. dernier a largement favorisé l'agrobusiness au détriment des petits paysans et de la transition vers une agriculture durable. Comme la plateforme, nous invitons le Gouvernement à faire de la PAC une véritable politique agricole et alimentaire commune. C'est l'occasion de réinsuffler des perspectives pour le secteur agricole secteur agricole français, tout en répondant aux fortes attentes de nos concitoyens, que ce soit en matière d'alimentation, d'environnement, de santé ou de lutte contre le changement climatique ! Monsieur le ministre d'État, merci d'avance de rassurer la représentation nationale quant à la triple ambition européenne, agricole et écologique de la France

que ce levier fantastique qu'est le budget de la politique agricole commune permette une mutation en profondeur de notre modèle agricole et, pour le dire de manière schématique, de passer d'une agriculture intensive en pesticides et à faible taux d'emplois ... Caricature ! ... à une agriculture intensive en emplois et à faible taux de pesticides. la politique agricole commune est une des plus anciennes politiques européennes ! Elle est nécessaire. Mais, vous l'avez dit, elle doit être adaptée aux enjeux et au contexte du XXI siècle. En ce moment même, Stéphane Travert est en train d'oeuvrer dans cette perspective à l'Assemblée nationale. Le premier axe-

nos exigences sociales et environnementales. La PAC doit donc contribuer à reconstruire cette fameuse indépendance alimentaire. Le deuxième axe de modernisation est la transformation de l'agriculture vers des modèles centrés, comme le demandent les consommateurs, sur la qualité, la réduction des pesticides et la protection de l'environnement. Ces services doivent être rémunérés ; ils doivent diversifier économiquement les revenus des agriculteurs. Par conséquent, la PAC ne peut plus être centrée uniquement sur les rendements. La course au « toujours plus » détruit en effet les fondements même de l'agriculture, c'est-à-dire les sols et leur biodiversité, ainsi que l'eau. Les aides doivent être dorénavant centrées sur ce nouveau modèle, à la fois protecteur pour la planète et les consommateurs

et républicain. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ils étaient quelques centaines, et ils sont maintenant près de 2000 à s'entasser au bord d'un canal dans les rues de Paris. Ce sont des migrants : ce sont des hommes, des femmes et, parfois, des enfants. Nous pouvons tous partager le constat qu'ils fuient une violence : la violence de la guerre pour certains ; la violence de la pauvreté pour d'autres. Ils fuient la violence d'une vie qu'ils jugent sans avenir. notre politique migratoire ne peut pas s'exonérer du respect des droits fondamentaux. Ces personnes doivent être mises à l'abri. Les élus du territoire, le maire d'arrondissement, la maire de Paris vous ont interpellé et vous ont adressé des propositions. Le Défenseur des droits s'est rendu sur place et a constaté des conditions de vie qu'il qualifie d'indignes. L'archevêque de Paris, Mgr Aupetit, est allé à la rencontre des migrants et a appelé à faire mieux ; il a parlé de « fraternité Quand allez-vous répondre autrement que par le silence à ces différentes interpellations ? Veuillez s'il vous plaît nous dire ce que vous comptez faire pour mettre fin à la situation de ce campement indigne. Bravo ! La parole

qui visait à réguler le flux de demandeurs d'asile en attente d'hébergement, est fermé depuis le 31 mars 2018, dans l'attente de la mise en place d'un nouveau dispositif composé de plusieurs centres d'accueil et d'examen des situations, ou CAES, en Île-de-France.

ma question porte sur la politique d'aménagement et d'équilibre des territoires. La semaine dernière, les trois principales associations d'élus locaux, représentant les régions, les départements et les communes, se sont exprimées conjointement pour dénoncer une « recentralisation du pays Nous sommes extrêmement attachés au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le plan Action coeur de ville et le futur plan d'action pour les hôpitaux sont des annonces positives. Toutefois, au-delà de telles mesures, les élus locaux assistent impuissants à la fermeture d'écoles, à la suppression des contrats aidés, au déclassement des zones défavorisées, à la détresse agricole, à la désertification médicale À cela s'ajoutent les menaces sur les petites lignes ferroviaires, ainsi que la dématérialisation des services publics, alors que le très haut débit n'est toujours pas dans nos campagnes. Tout cela intervient dans un contexte de baisse des dotations de l'État pour deux tiers des communes, soit 155 communes dans mon département. Les élus locaux et nos habitants sont inquiets. Il devient urgent d'adopter une vision nouvelle pour la ruralité et de mettre plus de cohérence dans l'action publique. Sans école, sans hôpital, sans justice, sans mode de transport, sans service public, sans internet, nos territoires ne pourront pas rester attractifs. Il faut donc une réponse globale qui touche tous ces secteurs en même temps. Il ne faut pas opposer le monde urbain au monde rural, mais tenir compte de l'équilibre des territoires et assurer l'égalité parfaite entre les citoyens. Le Gouvernement ne peut qu'être conscient de l'importance de la décentralisation. Je souhaiterais donc connaître ses intentions, monsieur le ministre de la cohésion des territoires. Quelles mesures concrètes pour empêcher la dévitalisation des territoires ruraux et assurer une cohérence indispensable entre ces différentes politiques

c'est le résultat- je l'ai déjà dit ici, et je le maintiens -de plusieurs décennies pendant lesquelles des fractures et des déséquilibres se sont malheureusement creusés de la République française. Nous en sommes tous responsables et tous conscients. Vous posez justement la question : comment pratiquer une politique de réparation ? Vous avez évoqué,

Dans mon département, comme dans les vôtres, la téléphonie fixe va moins bien aujourd'hui qu'il y a plusieurs années ; c'est une réalité ! Nous avons pris des mesures fortes

homogène sur l'ensemble du territoire de ce qui est prescrit au sein de l'éducation nationale grâce au Conseil des sages. Il s'agit donc d'un progrès très important. Vous en verrez les effets au fil du temps, selon les différents cas qui se présenteront. Je suis évidemment déterminé à faire respecter le principe de laïcité dans le système scolaire.

de février, dans la Nièvre, soixante-dix maires et adjoints ont remis leur démission pour protester contre la fermeture envisagée des urgences de nuit de Clamecy. À Saint-Claude, dans le Jura, c'est un bassin de vie de 60 000 personnes qui est privé de maternité et de chirurgie, au mépris de la loi Montagne ; celle-ci prévoit de garantir un accès terrestre aux soins dans des délais de transports acceptables. Madame la ministre, vos ARS amputent et stérilisent les territoires sans anesthésie. Démotivation des élus locaux certes, mais également de nos pompiers qui doivent assurer des transports de blessés de plus en plus longs. Ils sont à saturation du fait des innombrables sorties relevant d'un service ambulancier. d'incendie et de secours, les SDIS, paient des coûts de prises en charge pendant que l'État fait des économies. Les difficultés de gestion et d'organisation du système de santé ne datent pas de ce gouvernement, mais l'élaboration des projets régionaux de santé, les Les territoires ne peuvent pourtant pas se contenter de vous voir fermer maternités et hôpitaux en éloignant toujours plus le patient du traitement. Madame la ministre, allez-vous réviser les PRS élaborés de manière unilatérale et aujourd'hui rejetés ? Sinon, à quoi bon les soumettre au vote des assemblées locales ? La

Le ministère de la santé ne fait pas d'économies sur les territoires ; nous cherchons à les accompagner. Aujourd'hui, lorsqu'une maternité fonctionne avec des « mercenaires qui parfois ne sont pas présents, nous mettons en jeu la sécurité des patients. C'est le seul leitmotiv qui nous oblige quelquefois à fermer des structures, par manque de médecins disponibles sur le terrain. Les postes ne sont pas pourvus, vous le savez. C'est vrai pour les urgences et pour les maternités. C'est donc non pas une question budgétaire, mais une question de démographie. L'ARS cherche à accompagner les territoires dans un objectif de plus grande sécurité et de fluidité des parcours de soins. soins. Le PRS de Bourgogne-Franche-Comté, votre région, qui est très étendue, peu peuplée et qui fait face à de très grandes difficultés démographiques, tient compte de ces enjeux.

directeur général de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, Pierre Pribile, est tout à fait prêt à travailler de nouveau avec les collectivités. Aujourd'hui, l'enjeu sur les territoires est aussi un enjeu de sécurité pour nos concitoyens. Je rappelle que notre objectif prioritaire est d'assurer la qualité des soins partout en France, et j'y veillerai. Non, pas Madame la ministre, vous êtes ici dans l'assemblée des territoires. Auriez-vous besoin d'un ORL pour nous entendre ? Comme pour les enseignants ou les policiers, prenez les moyens d'affecter les médecins là où il y en a besoin, parce que, fermer les hôpitaux, cela ne supprime pas les patients ! La parole

le combat pour l'emploi est la priorité affichée du Gouvernement, notamment pour les publics qui en sont le plus éloignés. Le 4 avril dernier, vous avez choisi le Nord et l'hébergeur internet OVH pour lancer le volet numérique du plan d'investissement dans les compétences. L'objectif de ce plan est de consacrer 15 milliards d'euros à la formation de 1 million de jeunes peu qualifiés et de 1 million de demandeurs d'emploi de longue durée faiblement qualifiés, et de transformer en profondeur toute l'offre de formation. Les bénéficiaires seront à 80 % des personnes ne disposant pas du baccalauréat. Nous ne pouvons que nous féliciter que le Gouvernement intensifie et accélère l'effort de formation professionnelle des plus vulnérables pour les protéger contre le manque de compétences ou l'obsolescence rapide de celles-ci dans un contexte de bouleversements incessants du marché du travail. Vous l'avez répété dans le Nord, et nous partageons toutes et tous ici ce constat, personne n'est inemployable. Agir efficacement contre le chômage, c'est d'abord et avant tout développer les compétences, et chacun peut être ainsi formé aux métiers du numérique. Un jeune décrocheur ou une employée au chômage peuvent devenir codeur ou web rédactrice, car le numérique ouvre les portes et les ouvre grand pour les jeunes et les demandeurs d'emploi, quel que soit leur niveau de qualification. Lutter efficacement pour l'emploi, dans tous les secteurs, c'est l'affaire de tous : le Gouvernement, les régions, Pôle emploi, de nombreuses entreprises, en particulier les PME et TPE. Toujours dans le Nord, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, vous a présenté l'initiative Proch'Emploi, vise à aider les entreprises qui peinent à recruter à trouver plus rapidement leurs candidats à l'embauche. Cette initiative est née du constat que de nombreuses offres ne sont pas pourvues, alors que notre taux de chômage est très élevé. On voit bien, madame la ministre, et le dispositif des emplois francs que vous avez lancé officiellement cette semaine en est une bonne illustration, la nécessité d'une mobilisation générale et de la recherche de solutions toujours plus pragmatiques. Face à cette grande cause nationale, comment comptez-vous accompagner et encourager davantage encore le volontarisme des collectivités qui s'engagent résolument pour l'emploi ?

cette grande cause nationale de l'emploi, il faut que cela se fasse dans les deux sens. Vous avez rappelé l'initiative prise par Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, avec Pôle emploi, consistant à aller au-devant des petites et moyennes entreprises qui ne trouvent pas

socialiste et républicain. Ma question s'adresse à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice. Madame la ministre, vous présenterez demain en conseil des ministres un projet de réforme de la justice qui cristallise la colère des avocats, des magistrats et des greffiers. Ce projet éloignera encore un peu plus le citoyen de la justice, en portant atteinte au droit d'accès au juge. Par manque de lisibilité, vous laissez planer la suspicion sur la suppression du tribunal d'instance. est pourtant géographiquement proche des justiciables, simple dans son mode de saisine, financièrement abordable et parfaitement identifié par les Français, car il traite les litiges du quotidien. Vous prônez une justice dématérialisée, mais cette réforme aboutira à une justice déshumanisée. Vous ne prenez pas en compte la fracture numérique qui existe dans notre pays. Avec cette réforme, les victimes d'infractions devront déposer leurs plaintes en ligne, sans aucun accompagnement et avec des délais de réponse allongés.

La priorité est donc d'améliorer les moyens humains et financiers pour la rendre plus efficace. Il s'agit, et vous le savez, d'un souhait largement partagé au sein de cet hémicycle, car nous sommes tous attachés à la proximité des juridictions. Vous inquiétez le monde judiciaire par un manque de clarté, et les citoyens en portant atteinte à la justice de proximité. Pouvez-vous aujourd'hui, madame la ministre, devant la représentation nationale, clarifier la position du Gouvernement sur cette réforme ? La parole

je ne pense pas avoir à clarifier quelque chose qui me semble assez clair au regard de la multiplicité des occurrences au cours desquelles j'ai pu réaffirmer, ainsi que M. le Premier ministre, que nous ne fermerons aucun tribunal d'instance. Cela est très clair. Il y a plus de 300 tribunaux d'instance sur notre territoire, et tous, je dis bien tous, continueront

Dans tous les tribunaux, il y a des services d'accueil unique du justiciable qui sont implantés depuis un an : des personnes physiques accueilleront

que les moyens affectés à notre système judiciaire s'accroîtront de manière tout à fait importante. En cinq ans, 1,6 milliard d'euros supplémentaires et 6

le désordre règne à l'université. Des poubelles, des chaises, des tables sont transportées devant les portes d'entrée ; des cours et des examens sont suspendus. Le président de l'université de Lille m'a dit son inquiétude face aux pratiques des bloqueurs, notamment sur le site de la faculté de droit, de sciences politiques et sociales, que je connais particulièrement

Une note récente du renseignement territorial, dont vous avez certainement eu connaissance, indiquait : « Les blocages sont réalisés par une poignée de personnes qui n'ont, pour la plupart, aucun lien avec la sphère éducative. Quelques milliers face à 2,5 millions d'étudiants qui veulent travailler ! Il y a quelques semaines, le Président de la République souhaitait commémorer Mai 68. Il faut croire que les bloqueurs de facultés l'ont entendu, car ils sont en train d'exaucer son voeu. Pourtant, quelques jours plus tard, il dénonçait « les manipulations politiques extérieures responsables des violences dans plusieurs universités Alors, quel est le choix du Gouvernement ? Est-il bercé par la nostalgie de Mai 68 ? Comme à Notre-Dame-des-Landes, le rétablissement de l'État de droit se limitera-t-il au discours ? le Gouvernement est-il fermement décidé à user de son autorité pour qu'une minorité militante ne gâche pas l'année universitaire de la grande majorité des étudiants ? Où en êtes-vous, madame la ministre, et que comptez-vous faire pour que les étudiants puissent étudier ?

Lors de l'examen de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, vous avez rappelé à quel point vous étiez attachée à ce que les étudiants les plus défavorisés, les étudiants boursiers, puissent avoir accès à l'enseignement supérieur.

Élu des Ardennes, je peux en témoigner : le désarroi est devenu de la détresse. Les commerces disparaissent progressivement, mais comment gérer efficacement son activité quand on ne dispose pas du haut débit ? La fermeture des services publics se poursuit inexorablement. Le sud des Ardennes est en train de payer le lourd tribut de la carte scolaire. Des classes ferment, alors que les communes ont lourdement investi dans leurs écoles. Les élèves ont également des difficultés d'apprentissage. Ne méritent-ils pas, eux aussi, des classes à un seul niveau avec des petits effectifs ? L'accès aux soins est chaque jour un peu plus menacé. Ainsi, le centre hospitalier Bélair, à Charleville-Mézières, seul établissement de santé mentale des Ardennes, devrait subir une diminution une diminution des moyens accordés. S'ensuivra une baisse de la qualité des soins, qui ne permettront plus de répondre correctement aux besoins d'une population essentiellement rurale, sachant que la précarité frappe particulièrement les personnes en situation de fragilité psychique. Doit-on s'y résoudre ? L'abandon d'une partie de nos territoires est-il inéluctable ? La reprise en main des collectivités locales par la haute administration sera-t-elle sera-t-elle positive ? Monsieur le ministre, ces évolutions sont plus qu'inquiétantes. Entendez-vous la détresse des maires ruraux ? Qu'avez-vous à leur dire maintenant que vous avez quitté les travées du Sénat ? La parole est à M. le ministre de la cohésion des territoires. Monsieur le sénateur

qui nous propose un plan stratégique 2022 pour ce département. Il nous indique qu'il faut arrêter de consacrer des investissements publics à des sujets non prioritaires, et faire un audit sur ce qu'il serait particulièrement utile de développer en matière économique. Nous allons répondre

des collectivités, des élus, des forces vives de ces départements pour élaborer un plan constructif. C'est ce que nous allons faire ensemble, je vous l'assure

La séance est reprise. Nous reprenons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des données personnelles. Mes chers collègues, je vous rappelle que la discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte

non seulement aux présidents des assemblées, mais aussi aux présidents de groupes parlementaires. Cette mesure encombrerait notablement la CNIL, qui elle-même ne le souhaite pas et s'est montrée inquiète du risque que poseraient ses capacités de réponse dans ce cas-là.

ainsi que des personnalités désignées respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat qui siègent à la CNIL. Dans la rédaction actuelle du texte, les membres de la CNIL doivent en effet posséder une expertise large

L'Assemblée nationale a beaucoup hésité, en première lecture, puis en nouvelle lecture, sur le caractère alternatif ou cumulatif qu'elle souhaitait donner à ces deux compétences. Suivant la rapporteur, nos collègues députés ont finalement, après de nombreux doutes, adopté une disposition visant à rendre cumulatives les compétences exigées des cinq personnalités qualifiées membres de la CNIL. Il ne me semble pas inutile que les membres de cette autorité présentent des compétences dans chacun de ces deux domaines. Mais je comprends aussi la volonté d'élargir le vivier des candidats potentiels

le Gouvernement a été convaincu par l'argumentation présentée par la rapporteur du texte à l'Assemblée nationale : il lui a semblé opportun de renforcer la CNIL en termes de compétences aux techniques numériques, au vu de l'ampleur de ses futures missions. Pour ce motif, le Gouvernement a été défavorable à un amendement similaire qui a été débattu en séance publique à l'Assemblée nationale la semaine dernière. J'émets donc, à la suite de mon collègue secrétaire d'État chargé du numérique, un avis défavorable.

un jury qui représente, à parité, l'Assemblée nationale, le Sénat, les experts et les représentants d'ONG. Dans un souci de transparence, les auditions de ce jury seraient publiques et l'avis consultatif final sur les candidatures serait également rendu public.

M. Jérôme Durain. Le présent amendement a pour objet de rétablir la publicité de l'ordre du jour de la CNIL réunie en formation plénière, en renvoyant au décret le soin d'en définir les modalités. Il a pour origine un amendement déposé à l'Assemblée nationale. La publicité des travaux de la CNIL représente un premier pas vers davantage de transparence des travaux de l'autorité de contrôle, dont le rôle est appelé à croître eu égard à l'importance que prend la protection des données avec le règlement général sur la protection des données, prendre la forme de la télédiffusion de certaines délibérations de la CNIL, mais il existe de nombreuses autres modalités d'accès au travail de cette

Comme je l'avais expliqué en première lecture, la rédaction de l'amendement paraît beaucoup trop large, l'interdiction proposée risquant de paralyser l'activité des établissements dont la gestion des élèves et des notes est aujourd'hui très souvent dématérialisée. Si l'intention de départ est bonne, je ne peux souscrire à cet amendement,

parfois non pertinente pour certains traitements. En effet, le chiffrement n'est qu'une mesure de sécurité parmi d'autres, comme la « pseudonymisation ». Il ne peut donc pas être imposé systématiquement. Selon nous, il appartient aux responsables de traitement, au regard du principe de responsabilisation et sous le contrôle de la CNIL,

madame la ministre, mes chers collègues, je veux en préambule remercier fortement Sophie Joissains, notre rapporteur, de ses propos de ce matin,

automatiques mis en place dans les universités à partir des données collectées par Parcoursup. Ce corpus peut être soumis à différents traitements multiples sur lesquels nous désirons vivement, et je le souhaite comme vous, que la plus grande transparence soit faite. Il nous semble en effet, et c'est ce qui remonte du terrain, que certains critères ne correspondent pas à l'esprit de la loi, notamment le recours systématique à des tirages aléatoires, au tirage au sort. L'acharnement du Gouvernement à ne pas vouloir de transparence sur ces algorithmes locaux est destiné à cacher quelque chose qui commence à être avéré, c'est-à-dire le recours systématique au tirage au sort dans ces algorithmes mis au point au petit bonheur la chance par chacune des universités. J'aimerais, pour conclure, vous citer le propos de la rapporteur à l'Assemblée nationale : « Le Sénat a eu une position conservatrice peu compréhensible, visant à restreindre considérablement, et souvent en contradiction avec le règlement européen, le recours à ces outils d'aide à la décision. »

le fond les arguments de notre collègue Pierre Ouzoulias et de certains des membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. L'article 14 est, effectivement, d'une importance tout à fait considérable. Pour la première fois dans notre droit, il ouvre la voie à l'automatisation complète des décisions individuelles prises par l'administration. Je n'ai pas ménagé mes efforts pour convaincre nos collègues députés de la nécessité de trouver une rédaction de cet article protectrice des droits et libertés des citoyens. Le texte du Gouvernement ne comportait presque aucun garde-fou, et ceux qu'a ajoutés l'Assemblée nationale m'ont paru très insuffisants. Hélas, ces efforts ont été vains, car l'Assemblée nationale s'est pliée à la volonté du Gouvernement. Il en va de même du problème particulier de Parcoursup : les députés se sont contentés d'une demande de rapport au Comité éthique et scientifique chargé de superviser Parcoursup. Tout cela est désolant. Le rôle du Parlement n'est pas de demander des rapports, en même temps qu'il ouvre grand la voie à des dérives qu'il prétend dénoncer. Le rôle du Parlement est de fixer des normes et, en l'occurrence, d'obliger l'administration à respecter les droits des citoyens. qui concerne Parcoursup, je suis d'autant plus étonnée de voir le Gouvernement et l'Assemblée nationale rester sourds aux préoccupations exprimées par le Sénat que deux éléments nouveaux sont apparus depuis la première lecture. D'une part, dans sa délibération du 22 mars 2018 sur Parcoursup, la CNIL a relevé que la dérogation dont bénéficie Parcoursup aux règles de transparence prévues par le code des relations entre le public et l'administration était sans effet, sans effet, puisque la loi Informatique et libertés et le règlement européen lui-même comportent des règles similaires. Selon la CNIL, « les établissements d'enseignement supérieur qui recourraient à un traitement algorithmique pour examiner les candidatures qui leur sont soumises devront également fournir l'ensemble des éléments permettant de comprendre la logique qui sous-tend cet algorithme. » D'autre part, le Président de la République, dans son allocution du 28 mars 2018 au Collège de France sur l'intelligence artificielle, a clairement pris position pour la transparence dans l'usage des algorithmes, y compris pour l'accès à l'université. Il a d'ailleurs émis le souhait que des décisions ne soient jamais entièrement déléguées à un algorithme, ce qui va directement à l'encontre des dispositions prévues à cet article- il faut bien le dire. Pour le la clé est de mettre partout de la transparence publique sur les algorithmes, rendre les algorithmes publics, s'assurer qu'ils sont utilisés en transparence, traquer leurs biais, ne pas leur confier le monopole de la décision, s'engager à les enrichir ou les compléter par la décision humaine. » C'est ce que le Sénat avait prévu. ainsi : « Cette transparence, elle suppose une interaction permanente entre l'intelligence artificielle et l'humain et les choix qui seront faits, elle suppose des débats permanents, des corrections, elle suppose à partir du moment où on va mettre l'entrée à l'université, l'entrée dans une profession ou une formation derrière un algorithme, la nécessité de rendre plus démocratique cet algorithme et donc de s'assurer de sa loyauté, de s'assurer de sa transparence complète et qu'il puisse y avoir un débat sur ces règles sinon nous déléguons à l'algorithme le choix entre des priorités démocratiques.

Dans ce contexte, nous avons appris à la lecture du journal que l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche avait produit, à l'intention de la ministre de l'enseignement supérieur, une note de suivi particulièrement alarmiste. Dans cette note, l'Inspection générale aurait mis en garde contre un dispositif qui pose des difficultés philosophiques ou techniques liées à l'examen des candidatures. Elle aurait souligné que les établissements sont encore loin d'être prêts à examiner et à sélectionner les dossiers qui vont leur être soumis, que les critères appliqués varient d'une université à l'autre et sont parfois dénués de fondement légal. Bref, elle aurait déploré le manque d'accompagnement- c'est un minimum -du ministère.

souligner que le Gouvernement est extrêmement respectueux du bicamérisme, dans la manière dont il fonctionne sous la V République et tel que l'ensemble des articles de la Constitution l'a organisé-

Par ailleurs, au-delà des institutions, le Gouvernement est également extrêmement respectueux des femmes et des hommes qui composent nos deux assemblées.

en demandant à cette instance de rendre un rapport annuel sur les garanties de transparence de la procédure nationale de préinscription dans le premier cycle de l'enseignement supérieur.

la position de la commission pour que je ne renouvelle pas l'exposé très précis qu'elle nous a présenté précédemment. Je veux dire à quel point

Nous avons été sensibles aux informations de presse indiquant l'existence d'un rapport circonstancié de nature à confirmer nos inquiétudes. Oui ! Si je vous

mais vous savez à quel point le Sénat est attaché au renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement. Absolument ! Je crois d'ailleurs que ce parmi les intentions exprimées par le Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès, le 3 juillet dernier ; c'est un objectif auquel il attache lui-même de l'importance. Nous aussi ! C'est la raison pour laquelle nous attendons davantage de transparence de la part du Gouvernement. Cela dit, je suis prêt à saisir l'offre que vous nous avez faite de convoquer les responsables de l'Inspection qui ont approfondi ce dossier. Toutefois, je dois vous le dire, si leurs explications s'avéraient insuffisantes, nous reviendrions vers le Gouvernement pour, cette fois, non pas demander, mais exiger une information plus complète du Parlement. Je vous remercie par avance d'y être

rendre hommage à Mme la rapporteur, qui a fait le nécessaire pour que cet article soit révisé comme il se devait.

d'ailleurs l'objet de nombreuses contestations au sein des mouvements sociaux estudiantins, qui s'élèvent aujourd'hui contre l'exécutif- je reviens d'une manifestation où un certain nombre de groupes d'étudiants défilaient. Cette mesure n'est pas seulement injuste, elle est également illégale, puisqu'elle ferait exception

Cela n'empêche bien sûr pas de prôner la formation des plus faibles d'entre eux, de demander des moyens pour mieux les accueillir, d'accepter plus d'étudiants dans certaines formations sélectives, ni de mieux les former.

Malheureusement, il vous a un peu abandonnée ... Ensuite, de quoi parle-t-on quand on parle d'algorithmes locaux ? Je ne vous en donnerai qu'un exemple, celui du traitement permettant de pondérer les notes de contrôle continu en fonction du rang de classement des lycées.

je finirai mon propos en vous faisant remarquer que, bien évidemment, je connais le Comité éthique et scientifique. Figurez-vous que je l'ai saisi, voilà trois semaines,

sceaux ! Je ne souhaite pas répondre sur ce terrain, je vous dis ce qui est écrit dans les textes adoptés. Je tiens également à vous indiquer que le ministère de l'enseignement supérieur me fait savoir que les algorithmes seront effectivement publiés, sans doute au début du mois de septembre.

Ces amendements sont en partie satisfaits par le règlement général sur la protection des données. En effet, aux termes de l'article 8, paragraphe 1, du règlement, « lorsque l'enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n'est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant. » Or il est inutile et même interdit par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne de recopier ces dispositions dans le droit national. De plus, ces amendements visent à réintroduire une notion de double consentement qui n'est pas tout à fait convaincante, puisqu'elle conditionne la licéité du traitement des données des mineurs au consentement tant du représentant légal que du mineur concerné. D'un point de vue juridique, cet ajout ne semble pas compatible avec les termes du règlement, qui ne prévoit ni n'autorise une telle condition supplémentaire. En conséquence, je vous propose de nous en tenir au règlement général et sollicite le retrait

Ces amendements concernent la portée de l'action de groupe en réparation des préjudices matériels et moraux subis par les personnes concernées par la violation de leurs données personnelles, l'amendement n° 12 portant sur la date d'application de la mesure,

L'amendement n° 13 vise, quant à lui, à revenir sur le choix de la commission des lois de soumettre à un agrément de l'autorité administrative la faculté pour une association d'exercer une action de groupe en matière de données personnelles.

Nos collègues du groupe socialiste et républicain souhaitent que l'action de groupe en réparation des dommages dans le domaine des données personnelles entre immédiatement en vigueur. Ce n'est pas notre position. Par conséquent, la

L'agrément n'aurait pas été soumis à des conditions excessives, puisqu'il s'agissait simplement de s'assurer de l'activité effective de l'association, de la transparence de sa gestion, de sa représentativité et de son indépendance. Au reste, un tel agrément est requis en matière de consommation, d'environnement et de santé. Cela dit, le droit en vigueur comporte déjà de nombreux garde-fous, puisque seules peuvent agir les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et ayant pour objet statutaire la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel,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

Débat sur l'Union européenne face aux défis de la compétitivité, de l'innovation, du numérique et de l'intelligence artificielle. Personne ne